afin que les programmes scolaires comportent également des enseignements destinés à faire connaître la richesse de la culture et de la littérature francophones. La défense de la francophonie, vous le savez, est une priorité affichée par le Président de la République.

et notamment sa proposition n° 5, par laquelle nous formions le voeu d'intégrer les littératures francophones dans les programmes scolaires français. Notre pays accuse dans ce domaine un certain retard, contrairement à la Suisse, au Québec et à la Belgique, où la prise en compte de la francophonie dans les programmes scolaires fait l'objet d'une incitation claire. C'est pourquoi le livre blanc de la Fédération internationale des professeurs de français proposait également d'« ouvrir les curricula aux littératures francophones, aux différents patrimoines nationaux, aux variations linguistiques et culturelles, et plus largement à la francophonie ». Si, en 2015, le concept de « littératures francophones » a été introduit dans les programmes de français, les éditeurs de manuels scolaires n'ont pas encore emboîté le pas, et cette ouverture est restée lettre morte à ce stade. Or l'appropriation de la francophonie par la population française passera nécessairement par l'éducation et par la place qui est faite à la francophonie dans les programmes scolaires, présentation de la diversité des littératures francophones en cours de français et du monde francophone comme l'un des espaces de solidarité de la France dans le monde en cours d'histoire ou de géographie. C'est pourquoi je vous invite, mes chers

Rappelons cependant que l'Organisation internationale de la francophonie compte 88 États ou gouvernements membres, issus de cinq continents. Il y a bien entendu les pays d'Afrique francophone, mais aussi des pays comme le Qatar. chère collègue, me semble donc peu réaliste en termes de mise en oeuvre. Par ailleurs, sur le fond, il me paraît peu souhaitable de mettre sur le même plan l'enseignement des cultures de France et des outre-mer, d'une part, et de l'ensemble des cultures des nombreux pays de l'Organisation internationale de la francophonie, d'autre part. Enfin, le concept même de francophonie est largement au coeur des programmes d'histoire et géographie, aussi bien au collège qu'au lycée.

en puisant dans la littérature française, les littératures francophones et les littératures étrangères et régionales ». Il est également souligné que « les travaux portant [ ...] sur les littératures francophones montrent aux élèves qu'il existe des formules types d'expression française qui enrichissent par la création les pratiques du français.

je veux vous rassurer, l'enseignement moral et civique fait évidemment déjà largement référence à l'histoire de France, notamment en abordant les symboles de notre pays, ses institutions et ses valeurs.

Il requiert l'acquisition de connaissances et de compétences dans les quatre domaines de la culture civique et donne lieu à des traces écrites et à une évaluation. » Il y a donc clairement une explicitation de ce lien entre enseignement civique et moral. J'ajoute, et cela peut valoir pour d'autres

visant à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. C'est une excellente chose de faire connaître nos outre-mer dans le cadre de l'enseignement. Cela contribuera notamment à valoriser l'image de nos collectivités ultramarines, trop souvent mal perçues en métropole. Il faudra cependant former les enseignants à ces cultures. Pourriez-vous,

Il serait regrettable, en effet, qu'une mauvaise présentation des cultures d'outre-mer amène à enseigner des choses fausses ou mal expliquées. La parole

dans l'ensemble de la France renvoie à ce que nous disions hier sur la cartographie. J'ai pris des engagements clairs, dans la lignée de l'amendement présenté par M. Karam qui a été voté hier.

la connaissance des outre-mer fait partie de ces éléments. De même, notre formation outre-mer doit, elle-même, tirer parti de cette vision complète de l'enseignement.

: « Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. » Cependant, l'évocation de la France ultramarine dans les programmes scolaires est encore essentiellement réduite aux seules heures consacrées à l'étude historique des périodes colonialistes, esclavagistes et à l'étude géographique des zones économiques exclusives. La France ultramarine, dans sa diversité, représente près de 5 % de la population française. Sa richesse culturelle est l'héritage de décennies, de siècles de métissage sur chacun des bassins régionaux où elle est présente. Elle constitue 99 % du territoire maritime et plus de 80 % de la biodiversité de notre pays. Les outre-mer, ce sont des citoyens et des territoires français aux portes de la plupart des continents. Ils ont été, sont et seront plus encore les acteurs français d'enjeux majeurs pour l'avenir tant du monde que de la France. Une majorité des Français ignore cette diversité, cette richesse, dont elle fait pourtant partie. Cet amendement vise donc à ce que les élèves des DROM connaissent l'histoire de leurs territoires respectifs, qui se sont construits sur une agrégation de diversités culturelles.

des programmes d'histoire et de géographie dans les départements et régions d'outre-mer, afin de mieux prendre en compte la réalité historique et géographique de ces territoires. Par ailleurs,

? Monsieur le sénateur, je partage profondément l'esprit de votre proposition. Nous avons évidemment à agir dans ce sens. Comme vient de le dire le rapporteur,

des outre-mer, un certain nombre de progrès ont déjà été accomplis au cours des dernières années, voire des dernières décennies. Je l'ai d'ailleurs vécu moi-même lorsque, afin de prendre en compte les situations régionales particulières et les patrimoines culturels locaux, une pratique d'adaptation des programmes a été inaugurée dès 1999 dans les départements et régions d'outre-mer.

été concernés les programmes d'histoire et de géographie des cycles 3 et 4-du CM1 jusqu'à la troisième -, mais aussi, et pour la première fois, les programmes de sciences de la vie et de la Terre du cycle 4.

L'importance de certaines entreprises du domaine des nouvelles technologies montre à quel point le numérique est un secteur stratégique. L'apprentissage du codage informatique représente donc un enjeu majeur pour les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi. Pour notre pays, il s'agit d'un sujet crucial. En effet, la formation dès le plus jeune âge au langage informatique permettrait à la France de compter à l'avenir sur des ingénieurs suffisamment qualifiés pour s'assurer une indépendance numérique.

entrés en vigueur en 2016, prévoient, dès l'école primaire, une sensibilisation au codage informatique. Par ailleurs, il existe au collège un enseignement de l'informatique, qui comprend également le code, l'algorithmique et l'utilisation d'un traitement de texte.

de vote. J'insiste pour que l'on vote l'amendement de notre collègue Samia Ghali. La sensibilisation à l'informatique, la connaissance de l'informatique au sens large, cela n'est pas la même chose que la maîtrise du codage.

dire, cher collègue, être déconnecté et savoir gérer le codage, ce n'est pas du tout la même chose ! On peut tout à fait être déconnecté et apprendre le codage. Le codage, c'est le langage de demain. Autant nous expliquer qu'on n'a plus besoin d'apprendre à lire et à écrire parce que, de toute façon, demain, on saura tout faire avec des tablettes, qu'il suffira de parler et que les tablettes feront tout

pour mettre en oeuvre cette politique. Et cela n'enlève en rien au fond de ce qui a été dit, et que je partage totalement, sur les enjeux comme sur leur mise en oeuvre. On a ce que la loi dit et permet de faire. Il y a le plan d'accompagnement du ministre.

collège. Le sujet des écrans pose une question spécifique, qui n'englobe pas tous les sujets du numérique. Par exemple, la robotique, les enjeux de l'intelligence artificielle, qui sont sous-jacents, sont distincts

une culture informatique de nos élèves pour leur donner une capacité de maîtrise des outils et une aptitude à la distanciation. On peut, par exemple, apprendre le codage informatique sans ordinateur

que ce que nous venons de dire pour les élèves vaut,, pour les professeurs si on veut que tout cela se réalise. Il y a là, pour notre pays, un enjeu très important qui mérite le temps que nous venons de lui consacrer. Je voudrais non seulement vous rassurer, mais aussi vous dire que nous pouvons être vraiment à l'avant-garde sur ces questions.

faut anticiper ces évolutions. Cette précision sur le codage repose sur deux enjeux. La présidente Morin-Desailly et le ministre viennent de le dire, la question de la formation des enseignants est absolument

tout comme celle des adolescents, impliqués en permanence dans ce type d'activité. Il convient donc de permettre aux élèves, dès l'âge de 9 ans, de disposer des informations nécessaires pour maîtriser au mieux l'usage et les risques potentiels des réseaux sociaux. De nombreuses études préconisent d'ailleurs l'accès à internet sous contrôle parental à partir de l'âge de 9 ans. Il serait intelligent que l'école accompagne les parents et l'enfant au travers de cette démarche vers l'accès à ce nouvel outil dans ce monde immense et peu protégé qu'est internet. L'école doit donc participer à former des citoyens numériques avisés et responsables. Elle doit sensibiliser, au-delà de la manipulation, au discernement sur les réseaux sociaux afin de développer un regard critique. Cette information, cette acculturation, doit être graduelle. Commencer dès 9 ans, c'est permettre à l'enfant, tout au long des étapes qu'il va franchir dans la manipulation de cet outil et dans ce qui lui arrivera de la part de cet outil, d'être le mieux armé possible pour être en mesure d'y résister et de savoir l'utiliser.

l'heure ... L'article L. 312-9 prévoit qu'une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dès l'école élémentaire qu'elle comporte une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux sociaux. Dès lors, ajouter « dès 9 ans

Dans le cadre de cet enseignement, il est proposé de développer le travail de mémoire. Depuis 1961, le concours national de la Résistance et de la Déportation, le CNRD, s'inscrit dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et constitue une composante essentielle du parcours citoyen de l'élève. Les nouveaux programmes d'histoire du lycée ne prévoient plus l'enseignement des guerres du XX siècle en classe de première. Or cette année s'avère particulièrement adaptée pour permettre aux lycéens de participer activement au CNRD en mettant en oeuvre des projets collectifs. En supposant que l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale soit au programme de terminale, cela freinerait la participation des élèves déjà mobilisés par la préparation du baccalauréat. Alors que les actes antisémites commis en France ont progressé de 74 % en 2018, l'existence de ce concours doit plus que jamais être défendue, afin que les élèves perpétuent ce travail de mémoire de la Résistance et de la Déportation, source de leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui. Par cet amendement d'appel, vous l'aurez compris, monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur l'avenir du concours national de la Résistance et de la Déportation.

mémoire disparaissent, hélas, progressivement, c'est inévitable, ce concours, inscrit dans la durée et très au-delà des vies individuelles, est quelque chose d'essentiel pour la mémoire. Il durera, j'en suis certain, très longtemps puisque toute l'institution y est très attachée. Monsieur Grand,

toujours plus important du fait du développement des produits ultratransformés et tout emballés. Afin de lutter contre les risques sanitaires liés à l'alimentation, il est nécessaire de sensibiliser les élèves aux risques sanitaires et environnementaux qui découlent de la consommation d'aliments transformés et des emballages des denrées alimentaires. Les risques des produits alimentaires transformés ont notamment été mis en exergue

cours des dernières décennies, les habitudes alimentaires ont beaucoup évolué. Les Français consomment des produits ultratransformés : ces derniers représentent plus d'un tiers des aliments consommés. Il apparaît donc évident que l'éducation liée à l'alimentation doit prendre en compte les dernières recherches sur ces produits, afin d'inciter à un changement des habitudes alimentaires et de prévenir le risque de maladies liées à la consommation desdits aliments.

plus larges, tels que l'organisation des cantines ou l'éducation au goût, sujets eux aussi très légitimes. Pour ma part, je parle non plus d'éducation artistique et culturelle, mais d'éducation artistique, culturelle et sensorielle,

parole est à M. Jean-François Longeot. L'éducation au développement durable constitue une dimension essentielle de la transition écologique ; elle favorise, dès le plus jeune âge, les comportements vertueux et respectueux de l'environnement. Cette sensibilisation est d'autant plus importante que les jeunes influencent bien souvent les comportements de leurs aînés et contribuent, plus globalement, à enrichir la connaissance de chacun dans des domaines très variés, les enjeux environnementaux étant par nature transversaux. L'Organisation des Nations unies a identifié en 2015 l'éducation au développement comme l'un des dix-sept objectifs de développement durable. Dès 2013, sur l'initiative du Sénat, elle a été inscrite parmi les missions de l'école par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

Il vise à rendre cette sensibilisation plus pratique ; ainsi, les enfants deviendront des acteurs de la transition écologique. Par ailleurs, si l'éducation au développement durable constitue formellement l'une des missions de l'école, sa mise en oeuvre reste insuffisante.

Force est de constater que, selon les derniers indicateurs publiés, qui datent de 2016, un peu moins de 11 000 établissements, sur plus de 60 000, proposent un projet spécifique sur le développement durable

d'être sensibilisés au gaspillage alimentaire et à l'alimentation locale et durable, ainsi qu'à ce qui fait la vie de la Terre.

La mobilisation internationale des lycéens au sein du mouvement Youth for Climate démontre une véritable attente des élèves et une volonté d'action immédiate et concrète en matière de transition écologique. De plus, le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services rendu public le 6 mai 2019, estime que l'humanité doit changer profondément sa manière d'exploiter la nature. Ce rapport, qui recense la disparition imminente de plus d'un million d'espèces animales et végétales, prouve à quel point il est nécessaire d'éduquer et de sensibiliser les citoyens de demain à la défense des écosystèmes. La notion d'« urgence d'agir » est donc essentielle pour réinventer profondément notre manière d'exploiter la nature et n'a de sens que si l'on prépare les générations futures à ces changements politiques, sociaux, économiques et technologiques majeurs. Vous l'avez dit, monsieur le ministre : les jeunes sont créatifs.

Or ce changement culturel passe aussi par l'école. C'est ce qui s'est passé pour le tri sélectif. Nous proposons donc de préciser les programmes environnementaux qui pourraient être enseignés, avec une attention toute particulière à la ressource en eau et à sa consommation sobre, problématiques qui pour certains territoires. Nous proposons également de compléter l'esprit de ces programmes scolaires par une sensibilisation à l'utilisation responsable de l'énergie, mais aussi à la préservation de l'environnement. L'amendement

M. Roland Courteau. L'objet de cet amendement est de parfaire l'éducation à l'environnement et au développement durable. Éveiller les enfants aux enjeux environnementaux, c'est aussi leur montrer les impacts sur la santé des êtres humains. il apparaît nécessaire que cet enseignement visant à éveiller les plus jeunes aux enjeux environnementaux les renseigne sur les enjeux de santé environnementale. En informant les élèves des risques que peuvent présenter les agents chimiques auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans un système de consommation de masse-

des comportements nocifs pour la santé et nous encourageons des comportements permettant de mieux protéger l'environnement Ces comportements ne peuvent être adoptés que si les élèves ont conscience des enjeux qu'ils représentent et que s'ils s'ils sont suffisamment informés des agents chimiques auxquels ils sont exposés en permanence. Afin de pouvoir se protéger des agents chimiques auxquels nous sommes quotidiennement exposés sans forcément en être conscients, il est nécessaire de pratiquer des attitudes préventives sans lesquelles nulle personne ne peut se prémunir des risques auxquels elle est exposée, souvent de façon contrainte

L'effondrement massif de la biodiversité sur Terre est une réalité, malheureusement de plus en plus visible pour chacun d'entre nous. Moins d'oiseaux, moins d'insectes, moins de vers de terre. Les effets du changement climatique s'imposent à nous : inondations, fonte des glaciers, sécheresses. Or la biodiversité, c'est la vie, tout simplement. C'est un vaste tissu d'interactions constantes entre les espèces, nous compris. Sans le maintien de la biodiversité, nous pourrions être confrontés à une crise alimentaire mondiale. Dans notre malheur, nous avons une chance inouïe : la nature possède une capacité de résilience extraordinaire, proprement incroyable, peu qu'on évite d'intervenir. Par ailleurs, je tiens à attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la France métropolitaine- j'insiste sur cette précision -possède la plus grande biodiversité d'Europe. Nulle part ailleurs, ni en Europe ni dans le monde, on ne peut observer, en parcourant un même département, autant de paysages variés et d'espèces endémiques. La France compte 5 000 espèces différentes de plantes, alors qu'il en existe moins de 3 000 en Grande-Bretagne et autour de 2 000 en Pologne. Sur les 114 espèces de libellules dénombrées en Europe, 100 sont présentes en France. Ce sont nos terroirs, nés de notre histoire

Il est de notre responsabilité que soit enseignée, dorénavant, cette spécificité française, afin que nos enfants connaissent les enjeux de la réalité de tous les mécanismes des écosystèmes. Les enfants, qui sont notre avenir, doivent maîtriser ces sujets afin de devenir des citoyens éclairés et

la création de jardins botaniques et potagers dans les écoles, mais cela est déjà possible, cela existe même souvent, cela est mis en oeuvre dans bien des écoles. Rien aujourd'hui

vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

de notre ami Labbé. Cela me donne l'occasion d'émettre un avis, si je puis dire, sur les débats très importants que nous avons depuis le début de l'après-midi. Je pense, cher collègue breton, que votre appel à la sensibilisation et à l'éducation au développement durable est essentiel. Nul ne peut le nier. Toutefois, il me semble que l'amendement de notre collègue Maurey, défendu par M. Longeot, y répond. D'une manière générale,

avec l'État doivent, tout en conservant leur caractère propre, assurer un enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, doivent

avec l'obligation à laquelle sont soumis les établissements d'enseignement publics se justifie d'autant plus que les établissements privés sous contrat recevront de

par le biais de l'Insee, de collecter par bassin d'établissements des données propres à alléger le travail des professeurs et des parents. Une telle mesure de simplification administrative irait dans le bon sens et permettrait ensuite d'avoir une analyse fine du niveau de mixité sociale des établissements.

Aujourd'hui, seuls 29 % des Français seraient capables de maîtriser ces gestes, pourtant essentiels dans une situation d'urgence. En Allemagne, toute personne qui passe le permis de conduire est formée aux gestes de premier secours, mais une telle formation peut se faire beaucoup plus tôt. Cet amendement a pour finalité de permettre à chaque élève de quitter le système scolaire en étant titulaire du PSC1 afin de développer une culture du secourisme de masse, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays. Lors des débats à l'Assemblée nationale, le Gouvernement semblait favorable à cette idée, à condition de prévoir un délai suffisant pour mettre en place le dispositif et de former les enseignants.

Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation [ ...] aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité. Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. [ ...] « Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en

Or la perte de plusieurs semaines de scolarité est catastrophique pour ces enfants. Partir avant la fin de l'année scolaire implique en effet que le programme de l'année n'a pas été étudié dans son intégralité, tandis que revenir au-delà de la rentrée scolaire entraîne une réelle désorganisation dans la classe, les premiers jours de l'année scolaire étant déterminants pour tous les enfants. Leur intérêt implique par conséquent une scolarisation du premier au dernier jour de l'année scolaire. En outre, ces absences injustifiées constituent, il me semble, un manque de respect flagrant à l'égard des enseignants et de l'institution.

me paraît excessif, l'amende minimale pour un délit étant de 3 750 euros. Il me semble qu'une contravention suffirait. De plus, cet amendement pose un problème d'ordre constitutionnel,

Il n'est pas question de supprimer les allocations familiales, même si on pourrait dire, comme notre rapporteur, que l'absentéisme rejoint le manque d'assiduité dont nous parlions hier. Je vais donc vous donner la même réponse. Je pense que le contrat de responsabilité entre

pour savoir si le cours de maths ou de français sera assuré et qu'on leur répond que non, ils ont forcément tendance à garder leurs enfants à la maison ou à leur permettre d'aller se livrer à leurs loisirs.

Eustache-Brinio. La laïcité est un principe républicain auquel nous sommes très nombreux à être attachés. Il appartient aux élus de tous bords politiques de rappeler sans cesse qu'elle permet de lutter contre tout ce qui nous sépare et nous divise.

Le principe de laïcité doit être respecté et affirmé pendant ce temps scolaire. La sortie scolaire est un moment pédagogique qui s'inscrit pleinement dans le service public de l'éducation. Les personnes qui accompagnent les élèves lors des sorties scolaires, comme toutes celles qui concourent au service de l'éducation, deviennent des collaborateurs occasionnels du service public. Les personnes qui participent à des activités scolaires doivent faire preuve de neutralité dans l'expression de leurs convictions, notamment religieuses. Monsieur le ministre, vous avez vous-même rappelé ce principe et indiqué que vous considériez que le principe de laïcité avait vocation à s'appliquer au corps enseignant comme aux parents lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires. Un certain nombre de circulaires, au cours des dernières années,

sujet. Dans ces conditions, il est du rôle du législateur de clarifier les choses. Cet amendement a pour objet de faire appliquer le principe de laïcité partout où il doit l'être, partout de la même façon.

j'ai entendu bon nombre de sénateurs défendre la charte de la laïcité comme fondement de l'école républicaine. Je partage bien sûr cette position et je ne doute pas que ces mêmes sénateurs voteront cet amendement.

manifestant ostensiblement une appartenance religieuse aux sorties scolaires et aux personnes concourant au service public de l'éducation. Il vient clarifier utilement un flou juridique les jugements des tribunaux administratifs, l'avis de 2013 du Conseil d'État, les circulaires successives ont laissé les chefs d'établissement et les directeurs d'école ont laissé les chefs d'établissement et les directeurs d'école dans l'incertitude et font reposer sur eux la responsabilité de permettre ou non ces comportements. Comme le relevait le rapport de la commission d'enquête du Sénat de 2015, dont Jacques Grosperrin était le rapporteur, « la doctrine du " pas de vague " justifie des accommodements avec le principe de laïcité, faute d'une doctrine claire et opposable à tous les acteurs de la communauté éducative

de faire en sorte que nous prenions des mesures qui permettent de les régler efficacement et qui ne soient pas contre-productives. La parole est à Mme

Parce que l'école publique, l'école de la République à laquelle je crois, doit absolument rester laïque, je voterai cet amendement. La parole

somme toute assez claires en la matière, qui découlent de cette étude du Conseil d'État. Du reste, les arrêts des tribunaux administratifs sont conformes

J'ai longtemps pensé que les parents d'élèves pouvaient être considérés comme des collaborateurs bénévoles du service public, selon cette théorie qui veut que toute personne

Le scrutin est ouvert.

Le prosélytisme religieux, qui vise à convaincre une personne d'adhérer à une religion et n'est pas constitué par le simple port d'une tenue ou d'un signe religieux, est certes proscrit dans les services publics, mais il n'est pas interdit à la sortie des écoles, ce qui inquiète un certain nombre d'enseignants et de maires. Les

conserver un poids de santé, de réduire les risques de certaines maladies, mais aussi d'améliorer l'humeur et l'estime de soi, d'être en capacité d'obtenir de meilleurs résultats à l'école.

ans. Au titre de son rôle d'éducation et de santé publique, l'école doit permettre aux élèves d'avoir une activité physique suffisante et adaptée à leur âge. L'amendement

La jeune génération passe désormais plus de temps devant des écrans qu'en mouvement. C'est pourquoi la pratique des activités physiques et sportives doit être encouragée. Bien sûr, l'éducation physique et sportive, ou EPS, fait d'ores et déjà partie des programmes scolaires, mais l'objet de cet amendement est de rendre obligatoire, pour une durée minimale quotidienne, la pratique d'activités physiques et sportives, sans remettre en cause les heures d'EPS. Le jour où un cours d'EPS est prévu, cette pratique sera bien sûr considérée comme réalisée. Cet amendement se situe dans la droite ligne des objectifs du Gouvernement, monsieur le ministre : mise en place d'un label « Génération 2024 » dans les établissements scolaires ; volonté d'expérimenter dès la rentrée prochaine le projet « confiance et sport », avec classe le matin et sport l'après-midi.

des interventions auprès des écoliers et collégiens pour faire valoir la nécessité de pratiquer une activité physique régulière. Intervenir, c'est bien ; assurer une pratique, c'est mieux ! Ces activités physiques quotidiennes permettraient également de sensibiliser les jeunes générations aux valeurs du sport que sont le respect,

Toutefois, comme je l'ai expliqué en commission, il ne me paraît pas souhaitable de multiplier les injonctions à l'égard de l'école. Ce n'est pas au législateur de fixer l'organisation des emplois du temps et la répartition des horaires d'enseignement. prescrire des durées minimales reviendrait à figer l'emploi du temps des élèves, empêchant ainsi de prévoir des créneaux plus importants, nécessaires à la pratique de certaines activités comme la natation.

je demande le retrait de ces trois amendements. À défaut, l'avis sera défavorable.

de rappel d'un engagement de campagne du Président de la République, dont le programme électoral indiquait à juste titre que l'activité physique et sportive tout au long de la vie était un enjeu d'inclusion sociale, de développement personnel

enfants ont besoin de temps pour se construire ; étant moi-même maman d'un enfant de 3 ans, je peux témoigner que tous n'ont pas la même maturité. Cette mesure, vantée comme emblématique, permettrait nous dit-on d'améliorer l'apprentissage scolaire de l'enfant. Je ne partage pas cet avis. Aujourd'hui, 98,9 % des enfants âgés de 3 à 5 ans sont déjà scolarisés. Cette réforme ne concernerait donc que 26 000 enfants tout au plus.

La place médiocre occupée par la France dans les classements PISA doit nous amener à nous interroger ... Il est par ailleurs reconnu que l'avenir scolaire d'un enfant est quasiment scellé à son septième anniversaire, d'où l'importance capitale de conforter le premier cycle de sa vie scolaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle de mes voeux la mise en oeuvre de la scolarité obligatoire à 5 ans, afin de permettre la création d'un premier cycle dit « d'apprentissage des fondamentaux », intégrant la dernière année de maternelle, le cours préparatoire et la première année de cours élémentaire,

N'oublions pas, mes chers collègues, que ce chiffre est à mettre en perspective avec les disparités qui existent entre les territoires en matière de taux de scolarisation. J'entends les craintes de certains concernant l'augmentation des dépenses pour nos communes, qui devront s'adapter à la scolarisation des enfants D'autres déplorent un cadeau fait aux écoles privées. Sur ce point, rappelons qu'il s'agit d'abord d'une obligation constitutionnelle : l'État doit accompagner les communes lorsqu'il y a création d'une nouvelle compétence. Nous aurons l'occasion d'y revenir à propos de 4. Plus largement, je crois que les petites choses, les détails de mise en oeuvre ne doivent pas masquer l'objectif : l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire est une promesse républicaine que l'école doit tenir pour tous les Français. Je pense naturellement aux enfants de Guyane et de Mayotte, pour lesquels la scolarisation à 3 ans ne sera pas si évidente. Mais je pense aussi aux enfants vulnérables ou en situation de handicap.

À cet égard, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire est donc dans l'intérêt de la réussite de nos enfants, de tous les enfants. Mes chers collègues, voter en faveur de l'adoption de cette mesure, c'est voter en faveur de davantage de justice sociale et de l'égalité des chances pour chacun de nos enfants.

Dans les faits, de nombreux enfants sont déjà scolarisés dès 3 ou 4 ans sur mon territoire, où une organisation pédagogique, mise en place à la fin des années 1990, permet que l'enseignement en petite section se fasse dans la langue locale, avec une introduction progressive du français.

Si plus de 90 % des enfants ne maîtrisaient aucunement le français en 1996, ce pourcentage a bien évidemment baissé. Je sais que les responsables actuels du vice-rectorat et de l'enseignement privé sont ouverts à cette réflexion. Je sollicite votre soutien, monsieur le ministre.

nous pensons que, pour que ce soit un véritable progrès social, un progrès partagé qui suscite l'adhésion et la confiance, il faut au préalable répondre à quelques questions et apporter quelques compensations.

pour les communes et certains départements d'outre-mer. Nous y reviendrons ultérieurement. La scolarisation précoce des enfants répond à une préoccupation des sénateurs socialistes, qui, dès 2011, avaient déposé une proposition de loi visant à cette fin. Elle avait malheureusement été déclarée irrecevable

déjà présenté cet amendement. Cette mention aurait été inscrite dans la loi en 1881, époque à laquelle l'instruction des jeunes filles n'allait pas de soi. Si cette précision peut paraître aujourd'hui un peu surannée, elle nous semble toutefois constituer un gage contre toute éventuelle discrimination ou remise en cause des droits de telle ou telle catégorie d'enfants. À l'heure où certains droits des femmes qui paraissaient acquis sont remis en question, où les maires refusent parfois d'inscrire des enfants étrangers, primo-arrivants ou non, dans les écoles, pour des raisons souvent infondées, il nous semble important de maintenir cette précision. L'amendement n° 25 rectifié, présenté

concerne les enfants des deux sexes, français ou étrangers, avait du sens en 1881, tel n'est plus le cas aujourd'hui. La loi est très claire sur ce point : l'instruction obligatoire vaut pour tous les enfants,

la commission propose de ne pas remettre en cause ce qui constitue le coeur de ce projet de loi, à savoir l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction

trouvent pas complètement démunies en apprenant que leur enfant né en janvier ne pourra pas entrer à l'école.

particulier pour les enfants adoptés, afin de leur donner une réponse adaptée à leurs besoins. Le visage de l'adoption a considérablement changé ces derniers temps. Les enfants adoptés sont moins nombreux, mais plus âgés. Ils ont parfois

d'inscrire cette dérogation parmi les dispositions du code de l'éducation : un décret ou une circulaire suffirait, d'autant qu'il s'agit de décisions qui doivent être prises au cas par cas. D'ailleurs, des mesures adaptées sont déjà mises en oeuvre. La commission demande donc le retrait de ces amendements

J'ajoute que nous parlons d'instruction obligatoire, et non pas de scolarisation obligatoire. Autrement dit, un enfant adopté peut tout à fait, si l'adoption vient d'avoir lieu et si cela semble pertinent,

Ces dispositions seraient prises par les parents après avis consultatif du directeur de l'école. Quel est l'avis de la commission ? Mon cher collègue, vous savez très bien que le bon sens a été introduit par la commission à

désormais des dérogations à l'obligation d'assiduité en petite section de maternelle. Mon cher collègue, le bon sens que vous appelez de vos voeux est au rendez-vous grâce au travail de la commission,

à tous ceux qui n'ont pas encore tout à fait confiance en l'école maternelle, en sa capacité à donner aux enfants, en particulier aux plus défavorisés

24 élèves par classe, cela représente un seuil raisonnable pour améliorer les enseignements à ces âges et faciliter le travail d'acquisition pour tous, en tenant compte des divers degrés d'autonomie des enfants, et donc des contraintes s'imposant aux professeurs

de septembre 2021, le plafonnement des effectifs à l'école maternelle à 24 élèves par classe. Cet amendement a été victime de notre cher article 40

des demandes de scolarisation d'enfants de moins de 3 ans n'ayant pas abouti dans leur commune, pour transmission à l'autorité académique. La recherche a montré les effets positifs d'une scolarisation précoce, dès 2 ans, pour lutter contre les inégalités sociales à l'école.

: les parents ne sont pas tous hostiles à une scolarisation de leurs enfants dès l'âge de 2 ans, mais les écoles, faute de moyens et de personnel, accueillent de moins en moins les enfants de cette tranche d'âge. Nous défendons le droit à la scolarisation des enfants de 2 ans pour les parents qui la souhaitent, notamment dans la perspective d'un retour à l'emploi.